Cette baisse ne remet pas en cause le paiement des reliquats de droits ni le financement des investissements prévus par l'Agence

Selon les derniers chiffres du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, 718 000 étudiants perçoivent des bourses sur critères sociaux, soit 37 % des étudiants, mais 20 % d'entre eux vivaient malgré tout sous le seuil de pauvreté en 2019. Or la situation sociale,

financer le remplacement de l'indemnité inflation. L'adoption de cet amendement permettrait de ne pas remettre en cause l'objectif d'un soutien financier

de loi de finances rectificative et doté de 3,2 milliards d'euros, pour compenser l'ensemble des indemnités devant être versées ou remboursées par les organismes de sécurité sociale.

finances. Contrairement à l'indemnité inflation, la prime d'activité cible directement les travailleurs pauvres et modestes, qui sont les plus susceptibles d'être exposés

des publics. Les organismes qui versent le revenu principal vont être mis à contribution, dans un premier temps, pour mettre en oeuvre cette indemnité- employeurs privés, employeurs publics, Urssaf pour les indépendants,

l'emploi pour leur permettre de renforcer les aides à la mobilité qu'ils ont déjà la possibilité de verser au cas par cas aux chômeurs et jeunes en parcours d'insertion, notamment s'ils ont besoin d'effectuer des trajets en voiture dans le cadre de leur démarche de retour à l'emploi ». Ces aides devront donc être octroyées

doit se traiter dans la durée. Or ces aides, qui ne sont que ponctuelles, ne peuvent suffire à résoudre un problème de pouvoir d'achat qui s'inscrit dans la durée.

vous n'en restez pas là, puisque vous la remplacez par votre propre dispositif. C'est un cadeau électoral, qui, malheureusement, n'en est plus un, quand il est porté par le groupe Les

euros, bénéficiera de la prime de 150 euros. Une personne en couple avec deux enfants à charge, dont le conjoint est au SMIC, et gagnant entre 2 000 euros et 2 300 euros sera également bénéficiaire. Une personne en couple, avec deux enfants à charge et un conjoint sans ressources,

en considérant que les bénéficiaires de la prime d'activité sont les membres du ménage, alors que nous sommes sur une logique de calcul individuel de la prime. Même si nous ajoutons les bénéficiaires des minima sociaux, nous avons un désaccord sur ce chiffre. Au-delà,

combinée avec des mesures sur les tarifs, qui ont été évoquées, et avec un soutien spécifique des 5,8 millions de ménages les plus précaires ou les plus défavorisés, grâce à

Notre collègue propose d'abonder le programme « Soutien direct aux fédérations sportives » de 40 millions d'euros et de compenser par une majoration de l'annulation de crédits du programme « Sport » de 40 millions d'euros. Les dispositifs d'aide aux fédérations sportives existent dans la mission « Sport, jeunesse et vie associative ». C'est une solution pour aider les fédérations sportives, tout en préservant les finances publiques.

monsieur le ministre

propose de remplacer ce dispositif par un renforcement de 50 millions d'euros des moyens des opérateurs du service public de l'emploi au titre des subventions qu'ils ont déjà la possibilité de verser aux chômeurs et aux jeunes en parcours d'insertion.

l'accumulation des rapports n'est pas forcément le meilleur outil de contrôle pour notre assemblée. Quel est l'avis

1 946 014 ETPT sont matérialisés dans ce projet de loi de finances rectificative, par rapport au projet de loi de finances initiale,

de 226 ETPT. Au total, l'augmentation des emplois de l'État et de ses opérateurs s'élèverait à 1 106 équivalents temps plein travaillés. Trois missions sont fortement concernées : « Travail, emploi et insertion Solidarités et santé » et « Agriculture et alimentation ». Près du tiers de cette augmentation correspond à l'accompagnement de la réforme de l'organisation territoriale de l'État. Par ailleurs, 43 % de l'augmentation est liée à des renforts rendus nécessaires par la gestion de la crise sanitaire.

ces deux amendements. Ces deux amendements ont une logique commune. Régulièrement, on nous annonce qu'il faut réduire le nombre de fonctionnaires. On lance des chiffres à la volée, ce sont des dizaines de milliers de postes par-ci, des centaines de milliers de Puis, au rendez-vous de l'exercice du pouvoir, on se rend compte que les choses ne sont pas si faciles et on revoit à la baisse les projets de destruction du service public. Pour autant, même si,

Que voit-on en réalité ? L'État se désarme. Par ces deux amendements, qui sont des amendements d'appel- évidemment, nous ne souhaitons pas redistribuer les postes ! -, il s'agit de se donner les moyens de véritables politiques publiques ambitieuses

Dans une étude publiée au début de l'année 2021, le Centre d'observation de la société documente une évidence, à savoir que le taux d'épargne croît selon les revenus de la population. Ainsi, 40 % des Français épargnent en moyenne moins de 5

Exactement 40 160 foyers étaient concernés en 2018 par cette contribution exceptionnelle. Notre collègue Jean-Paul Dufrègne, à l'Assemblée nationale, nous apprend que le rendement de cette contribution s'élève à 1 milliard d'euros,

dans un esprit de justice fiscale, de demander un effort exceptionnel aux contribuables les plus aisés qui prendrait la forme d'un prélèvement assis sur le revenu fiscal de référence ».

est à M. Paul Toussaint Parigi. Le présent amendement vise à laisser aux services de la douane en Corse les compétences qui lui incombent en matière d'opérations liées à l'assiette et au contrôle du droit annuel de francisation et de navigation Rappelons, tout d'abord, que le présent article tend à prolonger un délai d'habilitation qui a expiré le 28 octobre dernier. Cela étant, son intention contrevient à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2022, qui prévoit l'abrogation du transfert du recouvrement de certaines impositions, dont le droit annuel de francisation, à compter du 1 janvier 2022. Par ailleurs, selon le rapport Gardette, les opérations liées à l'assiette et au contrôle du DAFN supposent l'expertise des « actes métiers douanes » qui ne sont pas transférables. pour le cas de la Corse, cette situation interroge sur le DAFN qui représente plus de 5 millions d'euros versés annuellement à la collectivité de Corse. Cet amendement vise à poser comme principe que la douane conserve la compétence pour le DAFN

? Comme vous l'avez rappelé, cet article 10 vise à proroger de deux mois et jusqu'au 31 décembre de cette année le délai de l'habilitation octroyé au Gouvernement par l'article 184 de la loi de finances pour 2020.

sur lesquelles le Conseil d'État sera amené à se prononcer, pour partie du moins. Une nouvelle habilitation pour vingt-quatre mois est demandée à l'article

Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement. J'ai eu l'occasion de préciser au président de la collectivité de Corse que le transfert du recouvrement du DAFN de la douane vers la DGFiP n'entraînera aucun changement sur les modalités de calcul du DAFN en Corse- elle connaît un abattement particulier -tant pour le montant payé par les contribuables que pour celui perçu par la collectivité. J'ai aussi échangé avec lui sur le devenir du bureau des douanes d'Ajaccio dont les effectifs vont être renforcés par rapport à ce qui était prévu initialement.

de 62 ans. Pour un salarié de moins de 62 ans, l'indemnité est assimilée à la compensation d'un préjudice. Elle est dès lors totalement exonérée. En revanche, les travailleurs âgés de 62 ans et plus ne bénéficient pas des mêmes modalités de rupture aux autres tranches d'âges. L'indemnité versée au salarié âgé de plus de 62 ans n'est pas soumise à une exonération fiscale. Cette disposition s'oppose aux incitations concernant le prolongement de la vie active

à ne pas être perdants sur toute la ligne.

: La parole est à M. Pierre Louault. La loi de finances pour 2021 a instauré un crédit d'impôt temporaire en faveur des PME pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments à usage tertiaire.

ce n'est pas seulement donner des objectifs de médailles, en distribuer au retour des jeux Olympiques et Paralympiques, organiser des soirées avec des sportifs à l'Élysée, dans le plus strict irrespect des règles sanitaires, règles sanitaires, ou jouer au foot et marquer un but devant un parterre de journalistes. Non, soutenir le sport, monsieur le ministre, c'est aussi tenir les engagements pris en direction du monde du sport ! Le 17 novembre 2020, soit il y a un an, jour pour jour, le président Macron s'est engagé à mettre en oeuvre une redevance d'image rénovée et applicable pour le sport professionnel. Vous-même, monsieur le ministre, vous étiez engagé, ici, dans cet hémicycle, à créer un groupe de travail. Ce groupe, qui a bien été constitué, a émis des propositions. Cet amendement vise uniquement, je tiens à le souligner, à réécrire le dispositif de 2017 qui ne fonctionne pas et est complètement inapplicable. Je connais d'ores et déjà vos arguments, monsieur le ministre, mais il ne s'agit pas d'une niche fiscale ni d'un quelconque cadeau, il s'agit d'une proposition concertée, acceptée par tous les acteurs dans le cadre d'un groupe de travail piloté par le cabinet de votre collègue ministre des sports. sports. Ce dispositif est avant tout voulu par tous les sportifs professionnels et vient uniquement simplifier le droit existant, à droit constant et dans la maîtrise des coûts.

Il serait un important que le Gouvernement passe des paroles aux actes, soyons ambitieux sur le sujet.

coûterait à peu près 50 millions d'euros. Il profiterait pour les trois quarts à des footballeurs qui gagnent plus de 13 000 euros par mois. Ce n'est pas tout à fait ce que j'entends par le soutien à l'émergence du sport professionnel ! Quant au soutien au sport,

Cette clause sera bornée dans le temps et subordonnée à des conditions proportionnées à l'objectif visé. Cet amendement s'inspire grandement de l'exemple italien.

Si l'entreprise a touché des financements publics, elle devra payer une amende. Pour revenir en France, nous ne pouvons pas permettre à des entreprises peu citoyennes- il y en a peu, mais elles existent

L'adoption d'une « clause anti-abus » aurait l'avantage d'apporter une réponse à ces cas concrets et de redonner un peu de force au discours du Gouvernement concernant la prévention des délocalisations.

Pour des groupes diversifiés, comment apprécier l'absence de délocalisation d'un site de production ? Permettez-moi d'élargir le sujet

La hausse des prix de l'énergie touche de très nombreux Français au pouvoir d'achat modeste ; cela nous rappelle l'épisode des « gilets jaunes ». En présentant une indemnité qui vise à compenser la hausse de l'inflation, le Gouvernement manque sa cible.

et par ce genre de mesures qui ne sont pas financées, alors qu'elles devraient l'être par une meilleure redistribution. Aussi, nous ne sommes d'accord ni avec

On continue la cavalerie financière ; pour faire face aux problèmes d'une génération, on reporte le coût sur les générations suivantes. Cela ne peut pas durer aussi longtemps que les contributions,

M. Michel Savin. Vous l'avez compris, mes amendements sont tous ciblés sur la politique du sport.

cet objectif de simplification semble être remis en cause par la diversité des revenus perçus par les sportifs non résidents, ce qui est difficilement compatible avec le système de retenue à la source.

L'adoption de cet amendement constituerait un acte de solidarité nationale fort, afin que nos collectivités puissent disposer de moyens supplémentaires pour développer des filières de recyclage et créer des emplois. Les élus locaux réunionnais sont unanimes pour demander à l'État de les soutenir dans cette politique ambitieuse et vertueuse. Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, votre votre position et votre vote sont déterminants pour ne pas entraver le nouvel essor de l'économie circulaire à La Réunion et ainsi faire du déchet une ressource. Quel

d'abord formuler un commentaire à l'attention de M. le rapporteur général. Si, chaque fois qu'un membre du Gouvernement participe à la pose d'une première pierre ou à une inauguration, cela se traduit par une évolution des dispositions fiscales, cela risque de me compliquer un peu la vie, en tout cas pour les fonctions que j'exerce

Il tend à une révision de la trajectoire d'augmentation de la TGAP pour La Réunion- hausse significative qui aura des conséquences à partir de cette année.

Les installations souterraines du laboratoire de recherche et du centre de stockage en couche géologique profonde de déchets nucléaires à haute activité et à vie longue sont développées dans la commune de Bure, située dans notre département.

et n'a que très peu de charges à transférer. Le solde est donc conservé par l'EPCI, qui regroupe 51 communes, 17 600 habitants, soit 336 habitants par commune en moyenne. Un tiers de ces communes bénéficient d'un accompagnement financier spécifique, une partie de leur territoire étant distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations de Bure- ce que l'on appelle la zone de proximité. De plus, la moitié de ces communes ont moins de 150 000 euros de recettes annuelles de fonctionnement. Mais force est de constater que, du fait de ce potentiel fiscal

à cette situation unique et catastrophique une correction dérogatoire, en excluant du calcul du potentiel fiscal des communes de ce groupement les bases de CFE localisées dans le périmètre de Bure. Je tiens à préciser que cette disposition ne concerne que ce territoire très spécifique de la communauté de communes des Portes de Meuse. Les adaptations visées par cet amendement sont liées au caractère unique du projet et sont sans conséquence pour le reste du territoire. Il s'agit donc d'un amendement très spécifique, important pour un territoire qui contribue

À ce jour, une dizaine d'athlètes paralympiques médaillés à Tokyo- dont toute la France a salué les exploits -sont touchés par ce problème.

L'article 90 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 prévoit que les primes « sont exclues des revenus pris en compte pour l'attribution des prestations en espèces ou en nature versées aux personnes du fait de leur handicap ». Malheureusement, monsieur le ministre, cet article non codifié est resté inappliqué et demeure méconnu. Par ailleurs, il est juridiquement peu opérant, selon les acteurs du mouvement sportif. Cet amendement a donc pour objet de codifier la loi de 2012 afin qu'elle soit accessible et utilisée.

Cependant, le texte est bloqué dans la navette parlementaire. C'est pourquoi il est urgent de faire adopter ce dispositif, qui touche peu d'athlètes paralympiques, mais peut les placer dans des situations difficiles. amendement vise à exclure les primes liées aux performances sportives du calcul des différentes prestations sociales versées aux personnes en situation de handicap.

sans avoir d'effets contraires. Il faut relever, en outre, que l'enjeu financier est mineur. Toutefois, si l'article 90 nécessite des précisions pour faciliter son application, il me paraît préférable de passer par la voie réglementaire.

de l'assiette de calcul de l'éligibilité à telle ou telle allocation. Tous les revenus sont pris en compte pour ce calcul, y compris les primes lorsqu'elles sont liées à des exploits sportifs. C'est une position constante du Gouvernement, depuis 2012.

notamment des entreprises de scierie, afin de sécuriser leur avenir. Il tend à une durée de provision de cinq ans au maximum, à échéance de laquelle, si aucune mobilisation n'est intervenue en investissement, les montants provisionnés sont réintégrés dans la fiscalité.

Quel est l'avis de la commission sur cette demande de coordination ?

vous ne semblez le dire ou le penser : souvenez-vous de la surprise qui a accueilli la montée de colère de l'automne 2018. Nous ne voterons donc pas ce collectif budgétaire, nous nous abstiendrons, parce que nous ne voulons pas non plus, à ce stade de l'année, voter contre

Tout d'abord, nous déplorons le manque de conditionnalité des multiples aides aux entreprises, lesquelles sont pérennes, elles. Ensuite, nous constatons que le déficit s'aggrave, mais que les plus aisés d'entre nous ne sont pas pour autant appelés à contribuer davantage.

Le scrutin est ouvert.